la C3S bénéficierait surtout au secteur financier, alors que la suppression de la CVAE pour la part régionale et de la CFE pour la part que nous diminuons

lorsque les entreprises ne sont plus à même de lutter contre la concurrence étrangère. Telles sont les deux raisons pour lesquelles le groupe Les Indépendants salue la baisse des impôts de production.

pérenne contre la concurrence internationale. Cet amendement se situe dans le prolongement de cette position : nous vous proposons d'aller au-delà et, comme l'a fort justement indiqué notre collègue Nathalie Goulet, d'intégrer

Une diminution excessive, à nos yeux, du taux de plafonnement remettrait donc en cause l'équilibre de la contribution économique territoriale, puisque, au lieu de limiter son montant lorsque celui-ci est trop élevé au regard de la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise,

est à M. Éric Bocquet. Par cet amendement, nous souhaitons limiter les conséquences négatives de la suppression de la part régionale de la CVAE. En effet, comme c'est le cas chaque fois que le Gouvernement s'attaque à la fiscalité locale- cela ne date pas d'hier -, des effets de bord ne sont pas anticipés et emportent des répercussions sérieuses au plan local. la suppression de la part régionale de CVAE, de très nombreux élus locaux ont alerté quant à ses conséquences sur le Fonds postal national de péréquation territoriale. Le contrat de présence postale, qui permet à La Poste de contribuer à l'aménagement et au développement du territoire de répondre aux besoins des populations, notamment des publics fragiles, est financé par ce fonds, lui-même alimenté par un abattement de taxe locale sur la CVAE. Le présent

des zones de montagne, des quartiers de la politique de la ville et des départements ultramarins, qui souffrent particulièrement, chacun le sait ici. Nous proposons donc, par cet amendement, de compenser la perte pour le Fonds postal national de péréquation territoriale afin que celui-ci soit au moins maintenu à son niveau de 2020.

d'euros, soit un gros tiers de sa recette. Comme je l'ai indiqué en réponse aux intervenants sur l'article, le Gouvernement travaille actuellement à une modalité de compensation ; nous sommes en discussions avec le groupe La Poste, en particulier, qui est directement concerné.

à cet amendement, c'est vraiment ne pas comprendre ce qui s'est passé ces derniers mois, et même ces dernières années, dans notre pays. La crise des services publics est vécue dans bien des territoires comme le symbole d'une forme de déclin du modèle français.

ne pas racheter d'actions et ne pas attribuer d'intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions

notamment pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extrafinancière. Les entreprises formalisent désormais une déclaration de performance extrafinancière, qui récapitule notamment les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique,

Les entreprises bénéficiaires de baisses d'impôt de production devraient ainsi, sous peine de sanctions, publier annuellement leur bilan carbone renforcé, qui doit permettre de suivre l'évolution des émissions directes et indirectes pour les postes d'émission significatifs, élaborer une stratégie interne de diminution des gaz à effet de serre, avec une trajectoire dès 2020 et jusqu'à l'horizon de 2030, ce qui rejoint la commande de la Convention citoyenne une récente demande du Conseil d'État. En outre, leur rapport devrait comprendre les plans d'investissements compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l'environnement et avec l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré.

Serait-ce même juste économiquement ? J'ai regardé : le non-respect des objectifs de l'accord de Paris pourrait coûter entre 115 000 milliards et 561 000 milliards d'euros,

et, en tout état de cause, que le moins de personnes possible soient victimes d'une perte d'emploi. Tel est le défi que doivent aujourd'hui relever les chefs d'entreprise.

tout cela allait créer des millions d'emplois et améliorer notre balance commerciale. Bilan des courses : c'est de moins en moins le cas.

M. Stéphane Artano. L'économie de la fonctionnalité privilégie l'usage d'un bien plutôt que son achat. Elle favorise une gestion optimale du cycle de vie des produits et participe à la préservation de nos ressources naturelles. Il s'agit ainsi de mettre un frein à la surproduction et à la surconsommation de biens en s'adaptant aux besoins réels des personnes, des entreprises, des collectivités et des territoires. Les entreprises ont un rôle important à jouer en matière d'économie circulaire, car leurs comportements sont de plus en plus vertueux. Il nous semble nécessaire de les accompagner par des mesures fiscales incitatives.

la définition de l'économie de la fonctionnalité retenue par ce bel organisme qu'est l'Ademe : « nouveau modèle économique [qui] constitue un véritable changement de culture consistant à sortir de la logique transactionnelle immédiate entre un fournisseur de produits et son client pour passer à un contrat de confiance évolutif et sur le plus long terme, nécessitant une véritable relation personnalisée et de proximité avec le bénéficiaire

la nécessité d'entériner une nouvelle dynamique de décentralisation afin de réinvestir les territoires ruraux en déclin. Le ministère de

au profit des jeunes pêcheurs artisans et des sociétés de pêche artisanale qui débutent dans la profession, et ce pendant les soixante mois consécutifs au lancement de l'activité. Face aux incertitudes qu'entraîne le Brexit et au risque de plus en plus grand d'exclusion des pêcheurs français des eaux britanniques, menaçant l'emploi et la cohésion territoriale des activités côtières françaises liées aux entreprises de pêche, il convient de protéger le premier maillon de l'industrie halieutique nationale en permettant aux armements de constituer des réserves financières.

au profit des artisans pêcheurs. Un tel dispositif permettrait à une entreprise de pêche artisanale imposée au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourraient être utilisées au titre de l'activité professionnelle au cours des dix années suivantes.

Par cet amendement, vous proposez d'étendre une disposition propre à la fiscalité agricole à un secteur qui relève d'une imposition au titre

avec pour mission de gérer des terrains et de les mettre à disposition dans le cadre de baux de longue durée, pour qu'on y construise des logements destinés aux ménages modestes, en accession ou en location.

une société anonyme (SA) qui revêt un caractère lucratif, en raison de sa forme juridique, est imposée à l'IS et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), quels que soient son objet et son activité, sauf dispositions légales contraires. En revanche, les organismes privés autres que les sociétés ne sont placés dans le champ de l'IS que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Ainsi, en application des principes dégagés par la jurisprudence, la détermination du caractère lucratif ou non d'un organisme sans but lucratif, repose sur une analyse au cas par cas. Il ne nous ne semble pas qu'une exonération générale soit le bon outil d'harmonisation.

pour les transactions immobilières qui concernent les logements dont la valeur est supérieure à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et l'application d'un prix de référence sur chaque territoire.

il ne lésera ni les grandes entreprises, ni les coopératives, ni les collectivités territoriales. Les entreprises unipersonnelles, généralement d'artisans, travaillent en nom propre

Les deux logiques sont clairement distinctes. Tout entrepreneur peut basculer vers le régime de l'EIRL et bénéficier à ce titre de l'option visée.

faut être précis. Un abattement de 6 000 euros du résultat imposable de l'impôt sur le revenu relève d'une logique totalement différente d'un taux réduit sur l'IS, puisqu'il peut aboutir à une exonération.

qui apporte, d'une part, des précisions sur les modalités d'application des correctifs portant sur les mécanismes liés à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, ainsi que sur les taux d'exonération et d'abattement de valeurs locatives afférant à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Il revalorise, d'autre part, les montants des seuils de revenus prévus pour l'octroi de dégrèvements de contribution à l'audiovisuel public en faveur des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans ou veuves, qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d'emploi ou disposant de faibles ressources. Enfin, cet amendement devenu l'article 42 a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle du code général des impôts sur les zones d'activités économiques. L'amendement que je présente aujourd'hui vise à insérer, en première partie

? Cet amendement prévoit que les dispositifs de correction, introduits par la loi de finances pour 2020, ne s'appliquent qu'aux impositions assises sur les bases communales et départementales de la taxe foncière. foncière. De plus, la suppression de la taxe d'habitation a eu pour conséquence d'organiser l'autonomisation de la contribution pour l'audiovisuel public et des allégements qui lui sont associés. En effet, jusqu'alors, cette taxe était assise. les seuils de revenus pour bénéficier du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public n'ont pas été actualisés pour 2021. Cet amendement prévoit donc de procéder à une actualisation, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre des bénéficiaires. bénéficiaires. Ces mesures auraient pu être anticipées davantage. Techniquement, le dispositif est calé et juste. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

que traverse notre pays, de nombreux producteurs de vins et spiritueux n'ont pu écouler leur production dans des conditions normales, et doivent ainsi faire face à une augmentation de stocks à la clôture de leur exercice entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021. Il est donc proposé un dispositif exceptionnel de déduction d'une fraction des charges de production du surstock, représentant 40 % de l'augmentation de valeur des stocks constatée entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, et plafonné à 40 000 euros.

? Cet amendement a pour objet d'augmenter les possibilités de déduction qu'offre le mécanisme de déduction pour épargne de précaution.

l'amendement n° I-75 rectifié. Pour faire face à la crise, les exploitants agricoles peuvent utiliser l'épargne de précaution constituée au cours des années antérieures, mais pour les seuls exercices clos à compter de 2020. Il est ainsi proposé de neutraliser les conséquences de l'utilisation de l'épargne de déduction pour aléas, et de déduction pour épargne de précaution sur le résultat fiscal réalisé en 2021, ainsi que sur le revenu professionnel de la même année, lequel doit servir d'assiette aux cotisations sociales agricoles. Par conséquent, ce dispositif exceptionnel et optionnel n'aura d'incidence que sur l'exercice de l'année 2021.

est l'avis du Gouvernement ? Cet amendement va au-delà de la jurisprudence du Conseil d'État, malgré la différence notable de situation entre la réduction partielle et totale du capital et en l'absence de rupture d'égalité entre les contribuables. Aujourd'hui, le choix qui s'offre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, savoir l'annulation partielle des titres ou la diminution de leur valeur, n'est commandé que par des considérations pratiques ou politiques de gouvernance de la société. Cet amendement créerait un biais fiscal important,

La crise sanitaire et les mesures de confinement renforcent un réflexe, d'ores et déjà courant en temps normal, des ménages : constituer une épargne de précaution. Il en résulte une épargne des Français abondante, mais insuffisamment fléchée vers des investissements productifs qui financent l'économie réelle sur le long terme. À l'heure actuelle, les PME, en particulier, ont besoin de financements en fonds propres pour innover et assurer leur développement. Les fonds d'investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) permettent aux particuliers d'investir dans les PME. Cet amendement vise donc à renforcer l'attractivité du dispositif IR-PME, en sortant la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement dans les PME du plafond de 10 000 euros. Il s'agit de créer un plafond spécifique

aux versements effectués tout au long de l'année 2020, ce qui, vous en conviendrez, ma chère collègue, constituerait un effet d'aubaine singulier pour les contribuables. Sur le fond, le plafond ne constitue pas, selon moi, le bon outil pour renforcer l'attractivité de cette réduction d'impôt, dès lors que tout excédent peut être reporté sur l'impôt sur le revenu au titre des cinq années suivantes.

puissent bénéficier de cette réduction d'impôt.

continue, pour 25 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales, elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Afin de permettre aux entreprises éligibles de continuer à attribuer des quel que soit leur mode de financement, une tolérance a été introduite dans les conditions d'éligibilité : il est permis aux sociétés cotées sur un marché réglementé d'attribuer des BSPCE à leurs salariés, dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, sous réserve que toutes les autres conditions de l'article 163 163 G du code général des impôts soient respectées. Le présent amendement vise à introduire une tolérance identique en étendant la dérogation, sous réserve d'un seuil de détention du capital de la société par des personnes physiques, directement ou indirectement,

Il faut savoir qu'une dérogation temporaire de trois ans est déjà prévue en cas de franchissement du seuil de capitalisation de 150 millions d'euros. L'amendement prévoit d'étendre cette dérogation aux conditions de détention

et ne respectant depuis plus deux ans ni la condition de détention par des personnes physiques ni le plafond de capitalisation boursière, à émettre des BSPCE, ce qui constituerait une dénaturation du dispositif. Par ailleurs, les entreprises ne pouvant plus émettre de BSPCE

Les 10 % les plus riches en ont même bénéficié de plus de la moitié : 54 % des 32 milliards d'euros de surcroît d'épargne.

dans cette situation de crise sanitaire, économique et sociale, à entendre de telles propositions d'amendements. Franchement, bravo !